Je suis la danse et je vous écris ; je suis la danse et je pleure ; je suis la danse et je meurs. » Madame la ministre, ce cri du coeur, exprimé cette semaine par l'interprofession de la danse, traduit un profond désarroi, partagé par l'ensemble du milieu culturel. Les artistes, privés de l'objet de la passion qui les anime et les fait vibrer, acceptent mal d'être frappés par des restrictions sans recevoir d'explications claires. Ce matin encore, le professeur Delfraissy refusait de justifier la mesure de fermeture des salles de spectacle ; le conseil scientifique rappelait en effet dans sa note préalable au deuxième confinement que « le risque de transmission est plus faible dans les théâtres et cinémas » que dans les autres lieux clos. Les artistes, coeur battant de notre exception culturelle, ne supportent plus d'être soumis à des dates couperets qui laissent entrevoir une reprise, avant de découvrir qu'il n'en est rien, pendant que d'autres secteurs reprennent leurs activités. Face à cette crise, nous avons salué la mobilisation de 2 milliards d'euros par le Gouvernement dans le plan de relance, même si nous regrettons que le crédit d'impôt au bénéfice du spectacle vivant, voté par le Sénat, ait été repoussé par l'Assemblée nationale. Pourtant, la réponse à ce grand vide ne saurait être uniquement budgétaire. Il faut rappeler avec force et passion que la culture n'est pas un secteur non essentiel. Au monde de la culture, le Sénat s'adresse clairement : le théâtre, le cinéma, les musées, l'opéra, les spectacles dans leur diversité sont essentiels, les artistes sont essentiels et nous avons besoin d'eux dans cette période de grande morosité. Puisque la culture est essentielle, je souhaite vous interroger sur deux points, Face à une interdiction généralisée, inadaptée et incomprise, ne faut-il pas étudier plus finement les règles d'ouverture des lieux culturels ? Quelles perspectives pouvez-vous proposer aux professionnels de la culture pour assurer une reprise sereine des saisons artistiques et de la visibilité dans leur programmation en 2021 ?

l'importance de la culture, qui est au coeur de notre projet politique, quelles que soient, par ailleurs, nos options idéologiques. Notre pays vit une tragédie avec cette pandémie, qui nous a imposé des sacrifices considérables dans tous les domaines et tout particulièrement dans le secteur de la culture, qui est le coeur vibrant de notre projet de société. Ce n'est pas de gaieté de coeur que nous avons adopté ces mesures de sécurité sanitaire. Je constate d'ailleurs que celles-ci sont partagées dans la plupart des pays d'Europe, que les lieux culturels sont fermés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, ainsi que- nous l'avons appris hier -aux Pays-Bas. Cela signifie bien qu'il y a un problème, une véritable crise sanitaire à laquelle il faut apporter des réponses adaptées. Nous avons été, nous sommes et nous continuerons à être, aux côtés de la culture. Vous préconisez des mesures sectorielles, celles-ci viendront sans doute, parce qu'il faut de la visibilité. J'y travaille avec les acteurs de la culture, que je rencontre de façon continue à mon ministère pour expliquer pour trouver des solutions. Nous en discutons aussi avec les parlementaires, en particulier avec les sénateurs. Le secteur a besoin de visibilité, nous aussi, mais ce temps n'est pas encore venu. Nous le préparons. Dès que nous pourrons desserrer l'étau sur le monde de la culture, nous le ferons. En attendant, nous l'accompagnons par des mesures financières fortes. Bien sûr, l'argent ne fait pas tout dans ce domaine, mais il va tout de même nous permettre de préserver l'outil culturel et d'accompagner ses acteurs, qui sont absolument indispensables à notre projet politique collectif.

EDF-GDF, c'était deux entreprises publiques qui disposaient d'un monopole ; EDF-GDF, c'était deux entreprises intégrées, de la production à la distribution, qui garantissaient l'accès à l'énergie partout sur le territoire un tarif réglementé ; EDF-GDF, c'était un savoir-faire des salariés envié et reconnu partout dans le monde ; EDF-GDF, c'était la souveraineté, l'indépendance et le patrimoine de la France. « C'était », car, depuis trente ans, les libéraux ont livré l'énergie au marché. Déréguler, déréglementer et privatiser, tel est votre seul credo. Les gouvernements successifs ont créé des acteurs alternatifs de toutes pièces, puis des mécanismes ubuesques, comme l'accès pour favoriser leur entrée sur le marché. Les résultats de la libéralisation sont les suivants : explosion du prix pour les usagers, devenus des clients, et dégradation des conditions de travail pour les salariés, devenus une variable d'ajustement. En moins de quinze ans, vous avez dépecé GDF, qui

Les deux premières, demandant le plus d'investissements, resteront publiques ; la verte, source de profits, sera privatisée. EDF sera ainsi privée de sa capacité à innover et donc à réussir la transition énergétique et écologique du XXI siècle. Plutôt que d'écouter la Commission européenne, qui vous demande de tout brader aux profits des intérêts financiers, entendez les usagers et les salariés mobilisés qui exigent un véritable service public pour défendre l'intérêt général. Madame la ministre, ma question est simple plutôt que d'organiser le black-out du service public, êtes-vous prête à renoncer à votre funeste projet ou à donner la parole au peuple français, par référendum, sur l'avenir de leur bien commun ?

le Premier ministre a pris hier, devant les députés, des engagements très clairs, que je veux réitérer devant vous. Comme vous le savez, la France a fait de la lutte contre le réchauffement climatique un axe essentiel de sa politique, en s'engageant sur l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans ce cadre, EDF joue et jouera un rôle capital dans notre pays, en étant l'un des principaux moteurs de sa transition énergétique. Pour réaliser nos ambitions, le Gouvernement, en lien étroit avec EDF, a donc engagé des discussions avec la Commission européenne afin de donner à cette entreprise les moyens d'assumer le rôle clé que nous souhaitons lui conférer. Il s'agit, tout d'abord, de mettre un terme au contentieux avec la Commission européenne, qui dure depuis plus de quinze ans, sur les concessions hydroélectriques, en permettant qu'EDF en conserve la gestion sans mise en concurrence. Il s'agit également de garantir le financement du parc nucléaire existant, en réformant la manière dont la production d'EDF est mise à disposition des fournisseurs d'électricité et,, est vendue à l'ensemble des consommateurs. Il s'agit de donner les moyens à notre pays de développer massivement les énergies renouvelables. Il s'agit, en outre, de préserver les consommateurs français contre les hausses de prix des marchés de l'électricité. Il s'agit, enfin, monsieur le sénateur, de conserver un groupe intégré dans lequel le statut des agents ne sera pas remis en cause. Vous le comprenez, nous ne souhaitons pas démanteler EDF, mais, au contraire, lui donner les moyens d'être un grand acteur, au niveau européen et mondial, de la transition énergétique.

le 18 novembre dernier, l'Organisation maritime internationale (OMI) a annoncé de nouvelles mesures en matière de décarbonation du secteur maritime. L'accord trouvé dans le cadre du 75 Comité de la protection du milieu marin porte sur deux points : mise en place d'une certification de l'efficacité énergétique, associée, notamment, à des mesures de limitation de la puissance des navires et instauration d'un système de mesures de l'intensité carbone. Ces avancées concrètes ont été saluées par la France, avec des réserves et une certaine prudence, d'abord parce que les propositions de la France et de l'Union européenne n'ont pas toutes été adoptées- c'est le cas, notamment, des mesures de coercition pour les navires les moins efficients ensuite, et surtout, parce que ces annonces ont un goût d'inachevé. Le secteur maritime, longtemps absent des négociations climatiques, est en effet responsable de 3 % des émissions mondiales de CO2. S'il s'agissait d'un État, il serait le sixième pollueur de la planète, loin devant la France et la Grande-Bretagne. Pire encore, l'accord obtenu à Londres ne devrait pas empêcher le transport maritime d'accroître ses émissions de gaz à effet de serre pendant la prochaine décennie, à rebours des objectifs de l'accord de Paris et de ses propres engagements, et alors que celles-ci n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Pendant ces négociations, certains ont accusé la France d'avoir revu ses ambitions à la baisse dans l'espoir d'obtenir un compromis, l'espoir d'obtenir un compromis, même fragile. Les prochaines négociations seront donc cruciales pour transformer les grandes déclarations d'intentions en réalités et nous savons pouvoir compter sur votre détermination ainsi que sur celle de la ministre de la mer. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser quel a été le rôle de la France au cours de ces négociations ? Que peut-on, par ailleurs, espérer des prochains cycles de négociation, notamment en ce qui concerne le financement de cette transition ?

c'est d'autant plus vrai pour des territoires comme le vôtre, pour lesquels le transport maritime est évidemment de première importance. C'est pourquoi, dans le cadre du plan de relance, nous déployons 200 millions d'euros

elle ne peut être présente aujourd'hui, car elle défend les intérêts de la pêche française à Bruxelles -pour obtenir des avancées concrètes. Vous l'avez dit, l'accord de novembre dernier à l'OMI comprend des avancées, mais il est imparfait ; toutefois, il s'agit d'un compromis, obtenu grâce à la mobilisation française dans un contexte international fortement dégradé. L'obtention de cet accord est une première victoire que nous devons saluer, prélude à de nouvelles négociations devant aboutir à de nouveaux engagements. Naturellement, nous ne nous arrêterons pas là : nous avons souligné, lors des négociations, notre souhait d'avancer sur l'instauration d'une mesure de tarification carbone sur les carburants marins ; nous participons aux travaux de réflexion sur l'extension du système d'échange de quotas carbone européen au transport maritime dans le cadre du Pacte vert pour ; nous soutenons, enfin, l'initiative de la Commission européenne, qui vise à développer les technologies bas-carbone. Je n'oublie pas l'importance de la mobilisation des parlementaires et de l'opinion publique sur ce sujet et je sais que je pourrai toujours compter sur la vôtre, monsieur le sénateur.

Avez-vous entendu le désarroi de ces professionnels du spectacle qui ne parviennent plus à suivre le fil de vos indécisions ? Le revirement des annonces du 10 décembre, avec, pour seul engagement à destination du monde de la culture, une date de revoyure, est le coup de grâce pour tout le secteur de l'activité culturelle nationale. La culture, qui pensait voir le bout du tunnel, replonge dans le noir. Le marasme de la politique que mène ce gouvernement est à la hauteur de l'incompréhension des acteurs culturels quand ceux-ci constatent l'affluence dans les grandes surfaces, dans les transports en commun ou dans les lieux de culte. La perspective du 7 janvier, à l'aube d'un possible rebond de l'épidémie, n'est pas plus rassurante. Alors, madame la ministre, comment comptez-vous faire pour que M. le Premier ministre lève immédiatement l'interdiction d'ouverture des lieux de spectacles vivants, en respectant, bien entendu, les règles sanitaires en vigueur ? Pourriez-vous indiquer clairement quelles sont les mesures envisagées pour préparer la relance en janvier, car rouvrir une salle de spectacle demande beaucoup de préparation Comment les acteurs culturels vont-ils être accompagnés dans cette démarche ? Quelles mesures concrètes et précises seront mises en place dès le début de 2021 grâce aux crédits du plan de relance que vous avez annoncé il y a quelques semaines ?

des différents opérateurs et acteurs de la culture, responsables de théâtres, de cinémas, comédiens ; nous sommes à leurs côtés. Je les entends, je les écoute

les conditions sanitaires. Le monde de la culture est extrêmement allant, il est prêt à s'engager, à réfléchir à la façon dont nous allons sortir de la crise, il est même prêt à faire des sacrifices supplémentaires sur les jauges, sur l'information, sur les différentes conditions sanitaires. Il nous faut également

Monsieur le Premier ministre, il ne suffit pas de mettre en place des protocoles sanitaires. Que faut-il pour que la culture redémarre et ne meure pas définitivement ?

vendredi s'est tenu une conférence ministérielle de la Grande Région sur le renforcement de la coopération transfrontalière dans le cadre de la pandémie. Les partenaires de la Grande Région ont été conviés, sur l'initiative de la ministre-présidente de la Sarre, pour signer une feuille de route de gestion de l'épidémie. Discuté depuis trois mois, ce protocole doit aboutir à une lutte coordonnée contre la crise sanitaire, sur des sujets aussi majeurs que la stratégie de dépistage et de vaccination, la prise en charge transfrontalière des patients, les secours d'urgence, la libre circulation, l'échange et le soutien matériel et humain, la mise en quarantaine ou encore l'échange de données et d'informations.

le Conseil européen de ce week-end a été l'occasion de traiter et de rappeler l'importance de ce sujet, mais, faute d'engagement concret de l'État, la déclinaison territoriale fait défaut. Comment expliquer, monsieur le ministre, que l'État n'ait pas signé un protocole de cette importance, alors que le Président de la République prône une Europe du quotidien et que ce sujet devrait être notre priorité absolue ?

Maurice Chapelan a écrit : « L'absence est un arsenic : un peu fortifie l'amour, beaucoup le tue », je me sens parfaitement fortifié avec vous aujourd'hui, et je constate que c'est réciproque. Je m'en réjouis ! Madame la sénatrice Guillotin, je vous remercie de votre question, qui m'offre l'occasion de rappeler que la France et le ministère de la santé sont pleinement engagés dans l'Europe de la santé. Vous avez raison, la pandémie de covid-19 a mis en évidence les limites de l'organisation de la gestion des crises par l'Union européenne, notamment le manque de coordination des États membres. Plusieurs initiatives ayant pour objectif d'améliorer notre préparation commune face aux pandémies ont néanmoins déjà été lancées. La Commission a ainsi présenté le programme renforcé, au sein duquel la résilience des systèmes de santé sera abordée ; elle a également annoncé une proposition législative visant à étendre le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), ainsi qu'une révision de la décision relative aux menaces transfrontalières graves pour la santé. Je m'en entretenais hier avec mes homologues allemand et portugais- le Portugal devant assurer la prochaine présidence de l'Union. La présidente de la Commission européenne a également annoncé un nouvel ensemble de mesures ayant pour objectif de renforcer

à l'esprit la mise en oeuvre d'une planification interrégionale de la préparation aux pandémies, qui reposerait sur la coordination des mesures sanitaires, l'identification et l'utilisation conjointe des infrastructures critiques situées de part et d'autre des frontières, la tenue d'un registre des capacités conjointes de réanimation ou encore la mise en place d'un système régional commun de transfert des patients et, enfin, le développement d'applications et de campagnes de communication multilingues dans les zones transfrontalières. La France est pleinement engagée, madame la sénatrice, dans le renforcement de l'Europe de la santé, j'y crois profondément, comme ministre chargé de ce secteur ; nous voulons une Union de la santé qui soit robuste, efficace, solidaire, cela constituera une priorité de la présidence de l'Union européenne que la France assurera à compter du 1 janvier 2022. La parole est Monsieur le ministre, nous sommes absolument d'accord sur les mots, toutefois je ne comprends toujours pas pourquoi ce protocole d'accord n'a pas été signé par la partie française. Dans le cadre de la présidence française de la Grande Région, qui débutera le 20 janvier, je vous convie à

Mme la ministre de la culture et concerne le maintien de la fermeture des lieux culturels. Madame la ministre, nous regrettons, d'abord, le manque de concertation avec les acteurs de la culture, y compris avec les collectivités locales, qui, comme nous, ont découvert ces mesures lors de l'allocution du Premier ministre, la semaine dernière. De plus, la transparence du processus décisionnel est plus que légère : annonces du Premier ministre le jeudi 10, suivies des recommandations du conseil scientifique le 12, puis de nouvelles annonces par le Premier ministre le 14, fondées sur ces recommandations, concernant, notamment, la présence des élèves en classe et l'autoconfinement. L'incertitude est ce qui pèse le plus sur les acteurs culturels. La CGT Spectacle appelle d'ailleurs à renforcer la commande publique culturelle dès maintenant, pour offrir aux professionnels une visibilité dont ils manquent cruellement aujourd'hui.

Théâtre, musée ou salles de concert favorisent pourtant un vivre ensemble qui resserre nos liens et répare les dégâts de l'isolement. La mise en balance des lieux pouvant ouvrir semble bien trop pencher vers les seuls commerces. Aussi, si le besoin de restreindre le brassage et la circulation des populations s'entend, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite savoir pourquoi vous n'envisagez pas d'opérer un rééquilibrage dans les décisions d'ouverture en faveur des lieux culturels, avec des protocoles sanitaires adaptés.

Cette visibilité, que demande à juste titre le monde de la culture, nous allons l'atteindre, nous y travaillons, parce que nous devons bâtir, avec les professionnels de la culture, un modèle résilient

Les universités sont parmi les derniers lieux à rester fermés lors de cette deuxième vague, avec les salles de théâtre, les cafés et restaurants, les cinémas et les salles de sport. Aussi saluons-nous l'annonce par le Gouvernement d'une reprise progressive, dès le 4 janvier, des cours en présentiel dans les universités. La vie étudiante devrait reprendre son cours, mais de nombreuses incertitudes subsistent. Nous disposons encore de peu de recul pour évaluer les conséquences de la scolarité à distance sur les résultats scolaires et le niveau des futurs diplômés, tous les étudiants n'ont pas accès à une connexion internet stable ou au matériel informatique nécessaire pour suivre les cours. Par ailleurs, le manque d'interactions sociales pèse sur leur quotidien, et peu d'étudiants bénéficient d'un accompagnement psychologique, la France ne disposant que d'un psychologue universitaire pour 30 000 étudiants. de nombreux jeunes s'interrogent sur la reconnaissance de leur diplôme par les professionnels, compte tenu des conditions actuelles d'apprentissage et des difficultés à accéder à un stage ou à une expérience à l'étranger. Madame la ministre, cette séance de questions d'actualité vient clore une année bien particulière

nous devons faire revenir les étudiants les plus fragiles au contact de leurs enseignants dans les universités. Je rappelle toutefois que les universités, pendant ce deuxième confinement, n'ont pas fermé

contre 6 % de leurs camarades de l'Union européenne ... Monsieur le ministre, vous occupez le fauteuil de Jules Ferry depuis trois ans et sept mois : vous êtes comptable, au moins pour partie, de ces résultats. Comment Comment expliquez-vous que se poursuive et s'amplifie cette trajectoire plongeante, qui inquiète les Français et fait mal à tous ceux qui aiment l'école de la République ?

Monsieur le ministre, vous m'avez répondu en fin connaisseur des rouages de votre ministère. C'est vrai, vous n'avez pas lésiné sur les réformes. Mais est-ce là vraiment le coeur du problème ? Au-delà des enquêtes et de leurs limites, la Nation constate chaque jour la baisse généralisée du niveau des élèves ; elle s'interroge et s'inquiète. Les mathématiques sont un révélateur implacable : elles ne font pas bon ménage avec une école qui freine les meilleurs pour que les autres suivent, une école qui a chassé de son vocabulaire les mots « effort », « notation », « mérite »

ne faut-il pas que l'école retrouve les chemins du dépassement de soi et de l'excellence ? Il fut un temps où un tiers des élèves de Polytechnique étaient d'origine populaire. Ils avaient rencontré des maîtres exigeants, qui ne leur parlaient pas d'inégalité de destin, mais d'effort et

il n'y a pas de deuxième session ! La parole est à Mme Michelle Meunier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

il apparaît que M. Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a délibérément influencé la rédaction du rapport de Santé publique France préconisant un stock de masques suffisant pour faire face à une pandémie. Monsieur le ministre, le fiasco des masques a profondément écorné la confiance de nos concitoyennes et concitoyens envers les décisions prises par votre ministère. Le fiasco des masques et la défiance qui s'en ont été le ferment de théories alternatives qui sapent le discours rationnel des décideurs. Le fiasco des masques a contribué à mettre en danger celles et ceux qui étaient en première ligne les soignantes et les personnels de l'aide à domicile, par exemple, longtemps démunis, mal protégés, potentiellement vecteurs de propagation et parfois eux-mêmes malades du covid-19. Ce fiasco des masques porte un nom : Jérôme Salomon. Monsieur le ministre, votre responsabilité politique est immense. À quelques jours du début de la campagne de vaccination, vous devez rétablir la confiance

Santé publique France a sollicité un comité d'experts, qui a répondu non seulement sur les antiviraux, mais aussi sur les antibiotiques, les masques, les respirateurs et d'autres produits. À cela, le directeur général de la santé a répondu, dans un mail de janvier également transmis aux sénateurs, mais non publié dans le rapport

commandé par Santé publique France a été publié en l'état ; son auteur, le professeur Stahl, un éminent infectiologue- grenoblois, ce qui ne gâte rien ... -, a reconnu lui-même qu'il n'avait pas changé un traître mot à son rapport et qu'il ne savait même pas de quoi il était question. Madame la sénatrice, je vous ai

le cap de la réussite pour la campagne vaccinale, il est encore temps de changer de capitaine

Les Républicains. Monsieur le ministre de l'intérieur, 132 agents sur 523 : ce chiffre effarant correspond au nombre de policiers de la circonscription de Grenoble qui ont adressé en début de semaine une demande de rupture conventionnelle de leur contrat de travail au préfet de l'Isère- de l'Isère- 25 % des effectifs ! À l'échelle du département, ils sont 180. Ce n'est pas tout : depuis lors, les policiers grenoblois assurent uniquement les interventions urgentes et nécessaires ; ils ont cessé toute patrouille, toute action d'initiative, tout contrôle. Cette situation n'est pas seulement inquiétante pour Grenoble, ville connue pour son haut niveau de délinquance et d'insécurité. Elle est inquiétante, car elle traduit un malaise profond et un véritable écoeurement de nos forces de l'ordre à l'échelle de tout le pays. Monsieur le ministre, les déclarations du Président de la République ont mis le feu aux poudres, lorsqu'il a validé l'expression « violences policières », parlé de « contrôles au faciès » quasi généralisés et annoncé la création d'une plateforme de dénonciation et de signalement. Avec ces propos, les policiers ont le sentiment d'être lâchés par le Président de la République ! Il est certain que des actes minoritaires, comme l'affaire Zecler, doivent être dénoncés et sévèrement punis. Mais, nous le savons tous, la quasi-totalité des membres des forces de l'ordre accomplissent un travail de très grande qualité. Pourtant, ces policiers qui assurent notre sécurité se sentent abandonnés. Pire, alors que leur mission est chaque jour plus complexe, ils subissent au quotidien des violences toujours plus nombreuses

a opté, en 2019, pour une stratégie de stockage hybride des données, consistant à recourir à de multiples hébergeurs. L'objectif est assez simple : garantir la réversibilité des choix de la banque publique, c'est-à-dire la possibilité de faire migrer ces données d'un hébergeur à un autre, sans être dépendante de l'un d'entre eux. Dans a noué trois contrats avec des fournisseurs de : Amazon, donc, mais aussi Microsoft et OVH. C'est dans ce cadre précis que Bpifrance a eu recours à la solution Amazon Web Services pour déployer, en cinq jours,

l'intégralité des données sont protégées par une clé privée, détenue et hébergée par Bpifrance, ce qui garantit la souveraineté sur ces informations. J'ajoute que la sécurité de la plateforme et du traitement des données a été d'ores et déjà contrôlée par l'Agence

Les administrations françaises vont-elles continuer à confier nos intérêts vitaux à des opérateurs extérieurs ? Prenons la mesure du problème et faisons confiance à des entreprises françaises ou européennes pour conserver

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. La date fatidique du 31 décembre 2020, qui marque la fin de la période de transition avant la mise en oeuvre du Brexit, approche. Londres va rompre ses dernières amarres avec l'Union européenne. En 2013, à des fins de politique intérieure, David Cameron, le Premier ministre britannique de l'époque, prenait le risque de proposer un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Proposer un référendum Depuis, Theresa May et Boris Johnson sont entrés dans une surenchère qui nous amène aujourd'hui à un divorce douloureux. Dès juin 2016, alors président de la commission de la pêche du Parlement européen, alerté la Commission européenne et les autorités françaises quant au risque que le secteur de la pêche soit considéré comme une variable d'ajustement d'un éventuel accord de sortie du Royaume-Uni. je n'ai eu de cesse de dire et de redire à mon ami Michel Barnier que ce risque devenait de plus en plus prégnant, et qu'il ne fallait pas dissocier l'accès aux eaux britanniques pour nos navires ni les possibilités de pêche du reste de l'accord, celui-ci devant être global. Aujourd'hui, nous nous dirigeons, au pire, vers un et, au mieux, vers un accord dramatique pour l'activité de la pêche en France. Ce secteur économique sera la première victime du Brexit. En effet, sans accès aux eaux britanniques ni aux quotas qui en découlent, de nombreuses entreprises des Hauts-de-France, de Normandie ou de Bretagne risquent soit de disparaître, soit de se rabattre sur d'autres zones de pêche, au risque d'épuiser la ressource. Le Premier ministre britannique a même fait sortir les navires de guerre de Sa Gracieuse Majesté. Ma question est donc simple, monsieur le ministre : que comptez-vous faire pour éviter ce désastre annoncé ? Quelles mesures allez-vous prendre pour éviter cette catastrophe économique qui paraît malheureusement inéluctable ?

La parole est à M. Joël Bigot, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre de la transition écologique sur la nouvelle prestation du Président de la République lundi devant la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention a formulé un ensemble de propositions pertinentes pour lutter contre le réchauffement climatique. Le groupe socialiste avait d'ailleurs fait siennes bon nombre de recommandations de la convention, qu'il a défendue lors de l'examen mais les quelques propositions qui ont eu la chance d'être adoptées par le Sénat ont été immédiatement effacées par les députés de la majorité gouvernementale. Ce matin, le Conseil national de la transition écologique

de l'obligation de rénovation énergétique, de l'écoconditionnalité des aides, de la végétalisation de l'alimentation, de la redevance sur les engrais azotés, du moratoire sur la 5G et j'en passe découle que le texte final ne comptera que 40 % des mesures recommandées par la Convention citoyenne pour le climat. C'est bien maigre, trop maigre au regard de l'urgence climatique. La crise sanitaire ne peut vous servir indéfiniment de parapluie pour dissimuler votre responsabilité dans l'échec de nos engagements bas-carbone. Le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat est sans concession : ce gouvernement n'a pas cessé de procrastiner et de reporter ce qu'il lui incombait de mettre en place, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Le Conseil d'État lui-même vous demande de justifier de votre inaction climatique depuis trois ans ! Et au niveau international, vous continuez à soutenir des projets gaziers et pétroliers jusqu'en 2035. Plutôt que de proposer à l'emporte-pièce un nouveau référendum opportuniste, soyez à la hauteur de vos promesses. Ma question est la suivante, madame la ministre : avez-vous l'intention de permettre un véritable débat démocratique en soumettant l'intégralité des propositions de la Convention au Parlement ?

un ensemble satisfaisant qui nous permette d'atteindre nos objectifs. Le Président de la République a d'ailleurs annoncé qu'il renforcerait les moyens du Haut Conseil pour le climat. Vous disposerez ainsi de tous les éléments pour qu'un vrai débat démocratique sur ces mesures emblématiques

mais nous voulons accompagner, aider le secteur à surmonter les difficultés. Vous avez cité les salles de cinéma. Je sais à quel point, au Sénat, vous êtes attachés à cet élément structurant des territoires, en particulier ruraux.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre de la transition écologique. Passionné de géographie ferroviaire, attaché au monde cheminot et au réseau ferré national- moins de 30 000 kilomètres de lignes sont ouverts à la circulation commerciale aujourd'hui -j'aurais volontiers posé des questions sur les trains d'équilibre du territoire, les trains régionaux, les lignes rurales ou le fret capillaire notamment, mais aussi sur les moyens humains auxquels nous sommes, comme vous, très attachés. Mais j'évoquerai dans ma question l'aménagement du territoire et les dessertes TGV, les lignes à grande vitesse

conseils généraux, les anciennes régions, les villes et les intercommunalités. Mais depuis la crise sanitaire- et même avant -, les extensions de desserte TGV sur ligne classique sont délaissées, abandonnées. Dans les Ardennes, la desserte s'arrête bien souvent à Reims-centre. Les villes de Rethel, Charleville-Mézières et Sedan ne sont donc pas desservies. Il en est de même pour des villes des départements de la Meuse, des Vosges,

le ferroviaire est une de nos priorités, comme en témoigne l'effort financier sans précédent que ce gouvernement a engagé en faveur de la SNCF : je pourrais citer les 35 milliards d'euros de dettes que nous avons repris, ou encore la recapitalisation à hauteur de 4 milliards d'euros que nous avons mise en oeuvre dans le cadre du plan de relance. Nous nous mobilisons aussi

Du fait du confinement et de la réduction des déplacements autorisés, les dessertes de certains de nos territoires ont fortement évolué ces dernières semaines : environ 30 % des TGV ont circulé et 60 % à 80 % des TER et ce, avec des horaires adaptés. Cela peut sembler faible, mais je tiens à préciser que la fréquentation était d'environ 10 % au niveau national et de 20 % en région Grand Est. Je rappelle aussi que la SNCF et ses salariés se sont mobilisés pour que ces déplacements se fassent dans de bonnes conditions sanitaires. Comme vous le savez, grâce au déconfinement, l'offre devrait atteindre près de 100

La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. En l'absence d'observations, je les considère comme adoptées.-

à ce qu'elle est issue d'une coopération renforcée entre vingt-deux pays. Le Sénat a toujours été très attaché à trouver des chemins intermédiaires

qui s'était faite la porte-parole des collectivités d'Île-de-France, en insistant sur la problématique des infractions dans les transports collectifs,

en compte un fonds spécifique de dotation, une gestion par la Caisse des dépôts et consignations, une cosignature du ministère de la justice et de Bercy, et enfin l'avis de l'Autorité de la concurrence.

la commission mixte paritaire a adopté hier, à l'unanimité, le projet de loi sur le Parquet européen et la justice pénale spécialisée. Les sujets abordés dans ce texte sont chers au ministère de la justice. Vous comprendrez donc le réel plaisir constater cette unanimité. Je tiens d'abord à saluer ma prédécesseure, Nicole Belloubet, qui avait engagé cette réforme auprès de vous, en février dernier. L'Europe et l'environnement, tels sont les deux thèmes qui ont été au coeur du texte et des débats. Cette loi prend date pour l'avenir, en permettant à notre institution judiciaire d'accueillir en son sein une structure innovante et opérationnelle, pour exercer directement l'action publique partout sur le territoire des vingt-deux États membres qui y participent. Le Sénat avait, il y a quelques années, émis un « carton jaune » pour s'opposer à la proposition de la Commission européenne créant le Parquet européen.

que le Sénat et d'autres parlements nationaux avaient émises, illustrant ainsi l'utilité de la procédure de consultation renforcée des parlements nationaux qui figure dans le traité de Lisbonne. Cette unanimité est aussi le fruit du travail réalisé sur un dossier qui, nous en sommes tous convaincus, devrait nous permettre d'être plus efficaces pour combattre les fraudes au budget de l'Union européenne. Les dispositions relatives à la justice pénale spécialisée améliorent significativement l'efficacité et la cohérence de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, la délinquance économique et financière.

ou les juridictions spécialisées, la justice sera mieux à même de répondre aux attentes de nos concitoyens en matière environnementale. Je suis heureux que le Sénat ait adopté ces dispositions audacieuses pour la justice environnementale et les ait complétées. Je pense notamment à la mesure permettant l'immobilisation d'un navire en cas de rejet des eaux de ballast par le capitaine. Ces ajouts, enrichis à l'Assemblée nationale par la création des officiers judiciaires de l'environnement, ont fait l'objet fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, et je m'en réjouis. Je remercie le Sénat, et en particulier son rapporteur Philippe Bonnecarrère, pour les diverses améliorations qu'il a pu apporter notamment aux dispositions du titre

mais surtout nous marquons ensemble le début d'une étape nouvelle de la construction européenne, celle d'une Europe qui dispose désormais de moyens renforcés pour faire respecter son droit. La parole

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le principal objet de ce texte est d'adapter le code de procédure pénale à la à la spécificité du travail des procureurs européens, délégués français nommés auprès du Parquet européen.

le projet a été présenté par la Commission européenne en janvier 2017, puis adopté par règlement, en octobre 2017, en Conseil « Justice et affaires intérieures

qui travailleront sur les sujets qui le concernent. En raison des spécificités du fonctionnement de notre justice, nous avons dû adapter le code de procédure pénale : les procureurs délégués pourront prendre des mesures qui relèvent normalement du juge d'instruction, comme les mises en examen. En revanche,

et le bon contrôle des fonds européens. En complément, le texte prévoit une spécialisation de la justice en matière d'environnement, afin d'améliorer le dispositif et de prendre en compte sa technicité. C'est une bonne initiative pour

puisqu'il s'agit de justice environnementale, pourriez-vous nous donner quelques éléments de calendrier sur la mise en place d'un délit d'écocide et sur le référendum constitutionnel qui vise à mieux intégrer la défense de la planète

le projet de loi que nous examinons comporte de nombreuses mesures et concerne de multiples champs de notre droit pénal. Le temps qui m'est alloué ne me permettra d'évoquer que certains de ces sujets, pourtant fondamentaux. À l'heure où le Conseil européen vient enfin d'adopter le budget et le plan de relance européens, l'importance du Parquet européen apparaît en pleine lumière. Son rôle est essentiel dans la lutte contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

La clarification que le projet de loi apporte au cadre procédural, à l'endroit des procureurs européens délégués, arrive au bon moment, pour l'entrée en fonction imminente du Parquet européen. Les deux assemblées ont pu apporter des précisions sur les compétences des procureurs européens délégués, notamment dans l'instruction et l'articulation avec les autres juges, particulièrement celui des libertés et de la détention. Nous serons vigilants aux premiers exercices des procureurs européens délégués et du Parquet européen. Je veux rappeler que ce parquet fait partie d'une construction plus large à laquelle Eurojust et Europol participent également. La coopération judiciaire et policière au niveau européen est essentielle pour la réussite de la lutte contre la fraude financière. Ce texte aborde aussi la question de la justice environnementale, qui a d'ailleurs fait son apparition dans le titre, lors de l'examen devant l'Assemblée nationale. Là encore, le dialogue entre les deux chambres sur des sujets d'intérêt commun aboutit à un travail équilibré. Cela permet de bien prendre en compte les diverses sensibilités qui demandent à s'exprimer sur les questions de justice environnementale. Il s'agit d'une base intéressante pour les travaux qui nous attendent durant l'année 2021. Nous serons amenés à nous prononcer, avant le peuple français, sur une intégration plus profonde des préoccupations liées à la préservation de l'environnement dans notre droit constitutionnel. Je tiens, à cette occasion, à rappeler notre attachement au bicamérisme et au rôle du Parlement dans l'élaboration des lois. Enfin, le dernier point que je souhaite aborder est la suppression de l'article 11 relatif à une nouvelle peine complémentaire, dite d'interdiction de paraître. Malgré les travaux du Sénat, qui avait tenté de rendre cette interdiction applicable, nous devons constater que l'instrument proposé n'était pas satisfaisant. La réflexion doit se poursuivre. Je souhaite que nous apportions des solutions adaptées au fléau des infractions graves,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, chaque année, on estime à plusieurs dizaines de milliards d'euros le préjudice causé à l'Union européenne par des actes de fraude et de corruption. Ces chiffres, gargantuesques, doivent nous interpeller sur l'urgente nécessité de renforcer la poursuite des auteurs de telles infractions financières, au niveau européen. C'est l'objet principal du texte sur lequel nous nous prononçons. Celui-ci vise, en l'espèce, à instituer un parquet européen, faisant ainsi droit à un souhait émis de longue date par la Commission européenne, ainsi que par certains États membres

d'autre part, l'amélioration des dispositifs actuels concernant la justice pénale spécialisée en France. Certaines de ces adaptations nous apparaissent particulièrement pertinentes et nous tenons à les saluer. L'instauration, en premier lieu, de pôles régionaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité environnementale est un nouveau concept intéressant. En effet, la multiplication des normes dans ce domaine en fait, à l'heure actuelle, un contentieux très technique. La spécialisation des magistrats est de ce fait une innovation positive. L'attribution, en second lieu, d'une compétence en matière d'affaires de pollution des eaux maritimes aux juridictions du littoral spécialisées est également une très belle avancée, que nous accueillons avec enthousiasme. Nous constatons la pertinence de ces adaptations, ainsi que, de manière plus large, l'importance de la création d'un parquet européen. sans moyens alloués à ces nouveaux pôles, sans formation concrète dispensée à ces magistrats, ces innovations risquent de souffrir des mêmes maux dont souffrent déjà les juridictions conventionnelles. En outre, l'article 8 interroge. Il tend à créer une convention, qui permettrait au procureur de conclure un accord avec une personne morale mise en cause pour un délit environnemental, en lieu et place d'un procès. Une telle procédure créerait une justice d'exception pour les délits environnementaux, en libérant les principaux pollueurs de toute reconnaissance de leur responsabilité. Allons-nous accepter que des délinquants environnementaux puissent bénéficier d'allégements procéduraux ? Allons-nous tolérer qu'ils puissent se soustraire à un procès public ? La protection environnementale n'est pas un sujet de second plan et ne peut, de ce fait, pâtir des complaisances d'une justice qui permet aux entreprises d'acheter leur impunité. Monsieur le ministre, mes chers collègues, si nous nous associons volontiers à l'objectif initial de ce texte, nous constatons que son manque d'ambition et sa faiblesse en matière de justice environnementale en diminuent grandement la visée.

Je ne peux que m'en réjouir car, compte tenu de l'ampleur des fraudes contre les intérêts financiers de l'Union européenne, il était indispensable de mettre rapidement en place un effort de répression concerté et conjoint. Nous espérions que ce Parquet européen soit opérationnel à la fin de 2020, mais la crise sanitaire qui a touché le monde entier nous a fait perdre presque une année, malgré l'engagement de la procédure accélérée en janvier 2019. La création d'un parquet européen, chargé d'enquêter et de poursuivre en justice les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, est un combat de longue date entrepris par la France, et une véritable révolution à laquelle ont pris part vingt-deux des L'adaptation de notre législation en ce sens représente donc une avancée majeure pour l'Europe. L'accord issu de nos travaux d'hier permettra également de renforcer la justice pénale spécialisée, notamment en matière d'atteintes à l'environnement, trop rarement poursuivies et sanctionnées. Un même mouvement a été introduit en matière civile par le Gouvernement en cours de navette. Ainsi, dans chacune des trente-six cours d'appel de notre pays, une juridiction spécialisée sur l'environnement sera créée afin de rendre des décisions civiles et pénales plus rapides et plus efficaces. La convention judiciaire environnementale permettra, quant à elle, une sanction plus rapide par le biais d'une amende, d'une remise en état ou d'une réparation du préjudice. Les conventions créées par la loi du 9 décembre 2016 relative à la Une peine pouvant atteindre 30 % du chiffre d'affaires et la possibilité de publicité de la convention seront, à n'en point douter, dissuasives. Le Parlement a opéré des apports importants en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. Je pense notamment à l'amendement permettant l'immobilisation d'un navire ayant jeté ses eaux de ballast dans les eaux territoriales. Je pense également à l'extension, sur l'initiative de nos collègues compétence des pôles spécialisés aux infractions ayant un fort impact environnemental, mais ne figurant pas dans le code de l'environnement. Cette nouvelle justice pour l'environnement va dans le bon sens, même si nous savons tous qu'il faudra aller plus loin dans le cadre d'une réglementation internationale. En dehors des mesures relatives à l'environnement, un certain nombre de dispositions ont contribué à enrichir le texte. Je citerai l'adaptation, proposée par mon groupe, du dispositif de spécialisation départementale des juridictions aux situations dans lesquelles le ressort d'une juridiction excède les limites départementales. Le Sénat a également enrichi les dispositions ayant tiré les conséquences de décisions du Conseil constitutionnel, relatives notamment à la possibilité de comparaître personnellement devant un juge en cas d'appel contre une décision de refus de mise en liberté ou en cas de saisine directe de la chambre de l'instruction, dans l'hypothèse où le JLD ou le juge d'instruction n'a pas statué dans les délais légaux. Je suis évidemment favorable à l'adaptation prévue à Mayotte de cette mesure, qui renforcera les droits des détenus, mais cela démontre, une fois de plus, les sérieuses difficultés qu'engendre le détachement de la cour d'appel à La Réunion. Voilà un exemple supplémentaire qui, je l'espère, monsieur le garde des sceaux, vous convaincra du bien-fondé de la création d'une cour d'appel de plein exercice dans le cent unième département. Je terminerai enfin en saluant l'entente à laquelle nous sommes parvenus s'agissant de la suppression de l'article 11, qui introduisait, dans le code des transports, une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun et dans les lieux destinés à leur accès.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, comme chacun sait, depuis 2016 et le référendum britannique, l'Europe subit malheureusement les rebondissements sans fin du Brexit. Les péripéties ont été nombreuses et n'ont pas toujours rendu service à ceux qui, comme au groupe du RDSE, défendent le projet d'une Europe mieux intégrée et plus vertueuse. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de poursuivre la discussion d'un texte participant au renforcement de la coopération européenne et à la mutualisation des efforts des nations qui la composent. De la même façon, nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur celui-ci, d'autant qu'il porte sur l'une des fonctions les plus fondamentales de nos pouvoirs publics. Sans en refaire l'historique, je rappellerai qu'il a été institué, en octobre 2017, au niveau européen, un parquet chargé de poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.

Plus particulièrement, comment se fera à terme l'articulation du procureur européen avec le juge d'instruction français ? Faudra-t-il de nouveau se poser la question de son existence ? Ces questions sont d'autant plus légitimes qu'elles ne concerneront qu'une minorité de pays au sein de l'Union européenne. D'où l'hypothèse que ces deux acteurs judiciaires peinent vite à accommoder leurs fonctions, puisque, du point de vue européen, nous voyons mal comment il pourra être tenu compte de ce binôme. Par ailleurs, le titre II du texte a pour objet d'améliorer la spécialisation de nos juridictions pénales. Sur ce point aussi, nous avons déjà fait certaines observations dont je redirai la teneur, car ce phénomène de spécialisation des juridictions pose mécaniquement le problème de l'accès à la justice. Des rapports et des avis nous alertent depuis longtemps à ce sujet la création de tribunaux spécialisés dans des domaines très limités peut conduire à une concentration de la spécialisation au sein d'un seul tribunal pour tout le pays ou pour une seule région. C'est évidemment un obstacle pour l'accès au juge, engendrant un risque d'éloigner le juge du justiciable, d'autant que l'accès à une justice dématérialisée de qualité, efficace et peu onéreuse demeure, malgré vos efforts, monsieur le garde des sceaux,

mise. Je terminerai en évoquant les dispositions du titre III, et nos regrets d'y trouver une forme de dispersion. Sans en contester le bien-fondé, il demeure que certaines de ces dispositions ne se rattachent ni à l'objectif d'instauration d'un parquet européen ni au renforcement des juridictions spécialisées. Sans doute n'y avait-il pas de wagon législatif plus pertinent, mais, comme toujours, nous nous méfions des textes balais et disparates, dans le détail desquels se nichent parfois de bien mauvaises surprises. Au regard de ces observations, le groupe du RDSE votera en faveur de ce texte.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, voté en début d'année par le Sénat, ce texte visait d'abord principalement à adapter notre organisation judiciaire et notre procédure pénale nationales à la mise en place, le 20 novembre, du Parquet européen. La réussite d'une telle mise en place pourrait être une belle démonstration de l'utilité de l'Union européenne, dans le contexte de crises politiques à répétition que nous connaissons. La lutte contre la criminalité financière semble en effet urgente à mener au regard des chiffres communiqués par la Commission européenne : la fraude transnationale engendre annuellement une perte de 50 milliards d'euros sur les recettes de TVA des États membres et les détournements de fonds européens atteignent 700 millions d'euros. Alors que l'accord sur le cadre financier pluriannuel à venir de l'Europe, ainsi que sur le plan de relance, a été conclu avec les plus grandes difficultés, il apparaît important de donner les moyens au Parquet européen de fonctionner, afin que les vingt-deux pays qui le composent avancent vers cet objectif commun sans discorde.

Mais, nous l'avons bien compris, le volet le plus emblématique de ce texte réside, paradoxalement, non pas dans son objet premier, mais dans le renforcement de la justice environnementale- point sur lequel nous restons pour Afin de remédier au très faible contentieux environnemental est instituée une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale. Passer par la justice dite « transactionnelle », d'inspiration américaine, ne nous laisse présager rien de bon sans la tenue d'un procès en bonne et due forme et avec des droits de la défense inexistants, ces conventions ne permettront pas une reconnaissance explicite de la culpabilité de l'auteur du délit. Et c'est sans parler des nouveaux pôles régionaux spécialisés, qui, en réalité, s'inséreront au sein des juridictions existantes et à moyens budgétaires constants. Pour notre part, nous considérons qu'il est urgent de créditer davantage la justice environnementale et, surtout, d'accorder de vrais moyens aux polices de l'environnement. Or force est de constater que les moyens des agences de l'État sont tous en rétraction, que ce soit ceux de l'Agence française pour la biodiversité ou ceux

nous saluons à ce titre la suppression par l'Assemblée nationale de l'article 11, qui instaurait une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun. S'agissant de l'introduction à l'Assemblée nationale d'un recours judiciaire possible

plusieurs orateurs l'ont déjà signalé, des milliards d'euros échappent chaque année à l'Union européenne et à ses États membres. Détournement de fonds européens, escroqueries aux subventions, corruption, blanchiment d'argent, abus de confiance, les causes sont multiples, mais la conséquence, elle, reste la même : une baisse des moyens alloués à la construction du projet européen. La fraude à la TVA intracommunautaire, cela a été dit, coûte à elle seule 50 milliards d'euros pour un budget de l'Union européenne de 148,2 milliards d'euros. La facilité avec laquelle on peut déplacer les capitaux dans le monde entier et la lenteur des enquêtes transnationales, qui se heurtent elles-mêmes à l'opacité de certains systèmes bancaires, pouvait, jusqu'à présent, que favoriser des vocations criminelles et force est de reconnaître qu'Europol, Eurojust ou l'Office européen de lutte contre la fraude n'ont pas su endiguer le phénomène. La création d'un parquet européen, chargé d'enquêter et de poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, sera, je l'espère, une réponse efficace. Cette réponse, nous la souhaitons, ici, au Sénat, depuis vingt ans bientôt ... En effet, dès 2002, notre assemblée adoptait une résolution appelant à la création d'un parquet européen. européen. Ce texte est donc un aboutissement pour nous, mais aussi un grand pas pour l'Union européenne. Bien plus qu'un agrégat économique, l'Europe se doit effectivement d'être porteuse de valeurs communes. Elle ne doit pas seulement être un marché intérieur ; elle doit être, aussi, une puissance qui nous protège et qui se protège. La formule retenue permet de garantir l'efficacité de la répression contre une délinquance astucieuse, largement internationale et dont les profits se chiffrent souvent en millions d'euros. Le texte qui revient devant notre assemblée aujourd'hui entend adapter la procédure pénale française aux règles de fonctionnements de ce nouveau parquet européen. C'est un travail bienvenu, qui permet de clarifier notre code tout en préservant ses spécificités, par exemple l'existence du juge d'instruction. En outre, et c'est aussi un point à saluer, ce projet de loi s'attache à muscler notre dispositif judiciaire face aux atteintes environnementales. L'attachement des Français à la biodiversité et au patrimoine écologique est sincère, le traitement des délits et crimes environnementaux est attendu et, d'ailleurs, si j'ai bien entendu les dernières déclarations du Président de la République, il est probable que nous débattions de nouveau de protection de l'environnement et de biodiversité dans les mois à venir. Le traitement des délits et crimes environnementaux, disais-je, est très attendu, car il n'est pas acceptable qu'il soit économiquement rentable pour une entreprise de causer un préjudice écologique ou de s'affranchir des règles permettant de préserver notre santé et notre cadre de vie. La création d'une sanction pouvant aller jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise coupable devrait être, enfin, dissuasive. Je pense aussi à nos élus locaux, trop souvent confrontés à des décharges sauvages, des permis de construire illégaux ou des infractions à la réglementation sur la pêche ou la chasse. L'État doit se tenir à leurs côtés, et c'est aussi le sens de ce texte.

ou encore la création d'une force de police, une sorte de FBI « à l'européenne », avec des pouvoirs d'enquête propre. Je soulignerai également le faible nombre de procureurs français délégués à ce parquet européen,

! Grâce à l'important travail réalisé par notre rapporteur Philippe Bonnecarrère, la commission mixte paritaire est parvenue à adopter un texte commun aux deux chambres. La création du Parquet européen est une bonne nouvelle. Alors que le Brexit évolue vers un épilogue douloureux, l'Europe réaffirme ici son souhait d'avancer dans sa construction, dans sa souveraineté et dans son identité. C'est donc une étape importante, historique même, en accord avec la conception que nous nous en faisons, entre respect de la souveraineté des États membres et coopération renforcée. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera ce texte.

Madame la présidente, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, comme chaque année, les délais d'examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture sont extrêmement serrés, et je n'ignore pas la difficulté qu'il y a à examiner un texte aussi volumineux

pour 2021, dans sa construction même, est un budget de soutien face à la crise sanitaire et de relance de l'économie. Il a été examiné dans un contexte particulièrement incertain, lequel explique l'importance des modifications qui ont été apportées au cours du débat. Afin d'éclairer la représentation nationale sur les conséquences de la crise sanitaire et dans le souci de sincérité qui anime le Gouvernement depuis le début de ce quinquennat pour chacun des documents budgétaires, je précise que nous avons été amenés à amender le contenu du projet de loi de finances chaque fois que nous disposions d'informations nouvelles

C'est ainsi que nous avons d'abord révisé, lors de la première lecture devant votre assemblée et en cohérence avec la loi de finances rectificative de fin d'année, le taux de croissance de-10 % à-11 %, le déficit public de 10,2 % à 11,3 % du PIB pour l'année 2020 et la croissance pour 2021 de +8 % à +6 %. Comme l'a souligné le Haut Conseil des finances publiques, ces nouvelles prévisions demeurent prudentes et nous l'assumons. Le passé très récent nous a montré qu'en matière de prévisions la prudence était certainement bonne conseillère. Afin de prévoir les nécessaires mesures de soutien en faveur des ménages et des entreprises en 2021 dans un contexte de prévalence épidémique, plusieurs dispositifs de la mission « Plan d'urgence

Tout d'abord, la dégradation anticipée de la situation économique en 2021 par rapport au texte initial du projet de loi de finances, de +8 % à +6 %, conduit à revoir à la baisse le niveau des prélèvements obligatoires pour un montant de 22 milliards Par ailleurs, le réarmement des dispositifs d'urgence porte ceux-ci à un niveau de 20 milliards d'euros l'an prochain, parmi lesquels 13,4 milliards d'euros n'étaient pas initialement budgétés.

d'autre part, un soutien des entreprises à hauteur de 8,6 milliards d'euros, dont 7 milliards d'euros pour le fonds de solidarité, 600 millions d'euros pour des secteurs particulièrement touchés par la crise- le sport, la culture et les stations de montagne -et 1 milliard d'euros d'aide au paiement des cotisations

l'accompagnement du groupe La Poste pour 66 millions d'euros : il s'agit d'assurer le même niveau de ressources au fonds postal national de péréquation territoriale, la réforme de la fiscalité locale que nous vous présentons diminuant mécaniquement cette ressource de 66 millions d'euros, que nous abondons par crédit budgétaire. Je pense aussi aux avances aux aéroports régionaux pour 250 millions d'euros, à la recapitalisation de l'Agence française de développement pour 500 millions d'euros, à l'achat de matériel sanitaire pour 430 millions d'euros et à une avance de trésorerie pour la campagne de l'aide alimentaire pour 120 millions d'euros. Nous avons, en outre, réévalué le montant du prélèvement sur recettes en faveur de l'Union européenne de 336 millions d'euros supplémentaires. Il s'agit là de la conséquence de l'adoption du cadre pluriannuel financier lors du Conseil européen de la semaine dernière. Ce Conseil a été marqué par cette réussite, qui permet la mise en oeuvre d'un plan de relance à l'échelon communautaire. Nous compensons les pertes de recettes du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » à hauteur de 300 millions d'euros et nous revoyons à la hausse, de 130 millions d'euros, notre estimation de dépense de l'allocation aux adultes handicapés

Les hypothèses macroéconomiques actualisées et les nouvelles mesures que je viens de vous détailler portent notre prévision de déficit public pour 2021 à 8,5 % du PIB, après un déficit de 11,3 % en 2020. Notre ratio d'endettement public s'établira à 122,4 % du PIB, contre 119,8 % en 2020. Il s'agit de niveaux jamais atteints, qui traduisent la violence de la crise que nous vivons.

et sur les restrictions aux secteurs économiques que celle-ci exigerait, y compris la prolongation de la fermeture de certains établissements recevant du public. Cette année un peu particulière n'a pas empêché des débats riches et fructueux au Parlement. Au Sénat, près de 600 amendements ont été adoptés en première lecture.

La lutte contre la pauvreté, ainsi que le soutien aux plus modestes, est une priorité et cette disposition participera à cette mobilisation. Le Sénat s'est également prononcé en faveur d'un amendement portant à 0 % le taux de TVA pour les vaccins contre la covid-19.

intercommunale (EPCI) auront l'assurance d'avoir, en 2021, au moins les mêmes recettes fiscales que le niveau moyen connu atteint entre 2017 et 2019, soit avant la crise sanitaire. De plus, la permission accordée aux administrations et aux établissements publics de donner leurs biens mobiliers aux fondations et aux collectivités territoriales a été confirmée en nouvelle lecture, tout comme l'harmonisation

Il se traduit, comme l'exercice 2020, par une dégradation des finances publiques à un niveau jamais atteint, qualifié d'historique. Nous assumons cette dégradation des finances publiques, dans la mesure où elle nous paraît constituer la seule réponse

à la situation d'un pays comme le nôtre, c'est-à-dire capable de faire face à ses engagements, de maîtriser son endettement et d'alléger le poids des prélèvements obligatoires sur la production de richesses nationales.

de continuer à échanger sur des textes budgétaires, ou d'autres textes relevant du périmètre de mon ministère, dans les semaines et les mois qui viennent. J'en suis ravi par avance. La parole

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie mercredi 9 décembre dernier, n'a pu aboutir favorablement, compte tenu de divergences trop importantes sur les 285 articles restant en discussion. En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient déjà adopté dans les mêmes termes 125 articles et supprimé l'article 19. À l'issue de la nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a parfois suivi, même le Sénat. J'en donnerai quelques exemples, avant d'indiquer les nombreux désaccords qui demeurent toutefois entre les deux assemblées. Parmi les principaux apports du Sénat qui ont été conservés par l'Assemblée nationale figurent tout d'abord les aménagements apportés au nouveau crédit d'impôt dont bénéficieront les bailleurs consentant des abandons de loyers à des entreprises particulièrement touchées par la crise, d'une part, en prévoyant son application dès l'imposition 2021, d'autre part, élargissant son périmètre notamment par la mise en place d'un mécanisme analogue de prise en charge partielle des abandons de loyers consentis par les collectivités territoriales. Ensuite, et c'est là probablement l'apport le plus substantiel du Sénat au projet de loi de finances pour 2021, l'Assemblée nationale a conservé le dispositif de l'article 22 B,

a également conservé, malgré un amendement de suppression de sa commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, l'article 43 C, qui prévoit la prorogation jusqu'en 2024 du crédit d'impôt cinématographique international.

postal national de péréquation territoriale, permettant ainsi de compenser les conséquences de la réforme des impôts de production sur ce fonds. plusieurs mesures de portée plus technique, de clarification ou de simplification de différents régimes juridiques, d'amélioration rédactionnelle ou encore de mise en cohérence avec le droit européen. Enfin, l'Assemblée nationale a suivi le Sénat sur la suppression de plusieurs rapports jugés inutiles. Pour autant, malgré ces apports du Sénat, des divergences importantes subsistent entre les deux assemblées et nombre des amendements adoptés par le Sénat, même lorsqu'ils ont été votés à une très grande majorité, voire à la quasi-unanimité, ont finalement été supprimés. ont finalement été supprimés. Le Sénat n'est pas toujours entendu comme il se doit ... Ainsi, d'un point de vue macroéconomique, il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas réalisé les efforts de maîtrise des dépenses publiques nécessaires pour redresser les comptes publics, alors que les indicateurs économiques du pays étaient encore « au vert » et afin que la France retrouve les marges de manoeuvre budgétaires utiles pour répondre le plus efficacement possible à toute crise, l'épidémie actuelle. Il ne faut pas perdre de vue l'impact qu'auront toutes nos décisions actuelles sur l'état de nos finances publiques à moyen terme. À ce titre, il aurait fallu privilégier des mesures temporaires, puissantes et bien ciblées, pour favoriser une sortie de crise rapide et dynamique. Concrètement, je le rappelle, l'État se finance désormais autant par l'endettement que par l'impôt. Si les taux remontaient, l'effort à fournir pourrait devenir insurmontable. plus, le plan de relance du Gouvernement est trop tardif, mal calibré et tient insuffisamment compte de la réalité vécue dans nos territoires. Ainsi, je regrette que l'Assemblée nationale soit revenue sur toutes les mesures adoptées par le Sénat pour que le plan de relance porte ses fruits à plus court terme. Il n'est qu'à citer le report en arrière des déficits dans la limite de 5 millions d'euros. Si le Sénat n'est pas revenu sur la réforme des impôts de production prévue par le projet de loi de finances, considérant que les entreprises, en particulier dans le secteur industriel, devaient voir leur niveau d'imposition se réduire pour que soit favorisée leur compétitivité, il importe aussi d'assurer une juste et pérenne compensation aux collectivités territoriales. Il est, à ce titre, très positif que l'Assemblée nationale l'ait suivi en conservant l'article 22 B. Toutefois, il est regrettable qu'elle n'ait pas conservé d'autres mesures retenues par le Sénat,

L'Assemblée nationale a aussi supprimé les deux contributions exceptionnelles adoptées par le Sénat visant, d'une part, les assureurs et, d'autre part, les grandes plateformes de la vente à distance, au nom de la solidarité nationale.

également dommage que la majorité gouvernementale ait refusé les dispositifs proposés par le Sénat pour renforcer l'aide à ceux qui se trouvent le plus en difficulté face à la crise, par exemple un fonds de solidarité renforcé visant à mieux couvrir les charges fixes ou l'aide à l'embauche. Du point de vue de la fiscalité écologique et énergétique, l'Assemblée nationale n'a pas suivi le Sénat qui préconisait un étalement sur cinq ans du malus automobile, accompagné d'un renforcement de la prime à la conversion. Cela aurait permis d'inciter davantage les automobilistes à faire le choix de solutions plus « vertes », sans tomber dans la fiscalité punitive. Je note que l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture certaines mesures auxquelles le Sénat s'était fermement opposé,

L'Assemblée nationale n'a pas non plus modifié les crédits des trois missions et des deux comptes d'affectation spéciale rejetés par le Sénat, de façon à faire évoluer la position de ce dernier. Enfin, le Gouvernement a fait voter par l'Assemblée nationale cette nuit, en nouvelle lecture, des mesures nouvelles loin d'être anodines. Certes, il est indispensable de soutenir les secteurs qui restent les plus durement affectés par la crise, comme les exploitants de remontées mécaniques des stations de ski ou certains acteurs de la culture.

prévoir que le programme 356 couvre non seulement les dispositifs de chômage partiel, mais aussi la prise en charge de congés payés de certains salariés et une aide exceptionnelle aux actifs permittents, saisonniers ou extras. En outre, plusieurs milliards d'euros de crédits ouverts en 2020 seront reportés sur l'année 2021, en particulier les 2,1 milliards d'euros ouverts sur le programme 356 par la quatrième loi de finances rectificative

mes chers collègues, les sujets de désaccords entre nos deux assemblées restent nombreux. Même si le Sénat proposait des modifications en nouvelle lecture,

le serait pour tout gouvernement ! Je tiens à cette occasion à vous remercier personnellement, monsieur le ministre, de nos échanges toujours positifs et constructifs tout au long des débats et de vos réponses toujours précises à nos questions.

pour la sortie du glyphosate, l'extension des exonérations fiscales et sociales en faveur des indépendants et de certaines professions libérales, l'extension temporaire du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs ultramarins, la prolongation de l'annulation de la taxe sur les spectacles due au Centre national de la musique Nous regrettons, en revanche, que d'autres dispositions votées par le Sénat n'aient pu être retenues. C'est le cas de l'article 54 relatif aux tarifs de rachat d'électricité produite par les centrales photovoltaïques. Son rétablissement pourrait avoir des conséquences lourdes pour un certain nombre d'exploitants agricoles liés à des opérateurs par le biais d'un bail à construction. Il faudra suivre ce sujet avec la plus grande attention. Concernant plus particulièrement les collectivités locales, je salue plusieurs avancées importantes intégrées à ce projet de loi de finances. Je pense au report de deux ans

En revanche, nous regrettons que notre proposition visant à engager le processus d'harmonisation des trois régimes de versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur Permettre de gagner une année afin de soutenir l'investissement local avait toute sa place et toute sa cohérence dans le plan de relance. De même manquent à l'appel la compensation de CVAE aux départements ou encore la compensation des pertes de recettes tarifaires des services

ouvre une perspective d'évolution qui, nous l'espérons, aboutira. Nous pensons également que d'autres avancées votées au Sénat pourraient être reprises à l'occasion du prochain projet de loi de finances Enfin, j'aimerais dire un mot sur la contribution des assureurs dans le contexte de la crise épidémique, sujet sur lequel le groupe Union Centriste s'est positionné très tôt, dès le mois d'avril dernier à l'occasion de Le Gouvernement n'a certes pas souhaité conserver le texte voté au Sénat, ce que nous regrettons. Néanmoins, grâce à ce vote, l'exécutif a pu disposer d'un utile instrument de négociation, les assureurs ayant finalement annoncé le gel des cotisations en 2021 pour les secteurs les plus durement affectés par la crise de la covid-19. C'est un premier pas. Pour conclure, compte tenu non seulement de l'échec de la commission mixte paritaire sur un grand nombre de sujets,

je vous remercie,

Je pense au crédit d'impôt incitant les bailleurs à abandonner les loyers au profit des entreprises locataires qui ont été les plus touchées par la crise, que l'Assemblée nationale a repris et élargi aux bailleurs sociaux, en en permettant une entrée en vigueur immédiate. Je pense également au maintien de la suspension du jour de carence pour les agents publics et au prolongement d'un an du dispositif Coluche pour les dons aux associations d'aide alimentaire. Je pense enfin aux avancées adoptées sur l'initiative de notre groupe, qu'il s'agisse de la TVA à 0 % sur les tests et vaccins contre la covid-19 du crédit d'impôt visant à accompagner les agriculteurs qui ont fait le choix de sortir du glyphosate. Ces mesures ont été retenues et enrichies par l'Assemblée nationale au cours d'une longue nuit de débat.

... En effet, et c'est presque devenu une habitude, en dépit de toutes ces avancées, nous aurons à discuter dans quelques minutes d'une motion tendant à opposer la question préalable. Projet de loi de finances pour 2018 : le gouvernement était tout juste nommé et les députés venaient à peine d'être élus que, déjà, le Sénat déposait et votait une telle motion. Projet de loi de finances pour 2019, premier budget de plein exercice de la nouvelle majorité présidentielle

que quatre plans d'urgence d'une ampleur inédite ont été mis en oeuvre, que l'État n'a jamais failli dans son soutien aux entreprises, aux collectivités, à nos concitoyens, et que nous, parlementaires, avons su

notamment les crédits nouveaux pour la culture et pour les remontées mécaniques, les 5,6 milliards d'euros pour le fonds de solidarité, les aides aux permittents, aux saisonniers ou aux extras -, jugeant

en contradiction avec ces avancées que beaucoup semblaient reconnaître, qu'une nouvelle navette parlementaire ne serait pas de nature à faire changer d'avis nos collègues députés. Je crois, pour ma part, que renoncer n'est pas le meilleur moyen d'y parvenir.

Les débats en nouvelle lecture auraient pu nous permettre d'y voir plus clair, de clarifier nos positions et d'ajuster ou de renforcer ce qui aurait pu l'être. Cette année encore

soulève, une nouvelle fois, la question de la capacité à légiférer correctement dans des conditions de travail aussi ubuesques, qui ne cessent de se dégrader d'année en année.

il reste un effet collatéral déjà observé ces trois dernières années : les articles non rattachés sont devenus une sorte de « troisième partie » du budget, avec plusieurs dizaines d'articles supplémentaires- et non des moindres, parfois ! -et des mesures comme la prorogation en 2021

il sera impératif de veiller strictement à la bonne exécution de ces crédits supplémentaires. Les Français ne croient plus à l'argent magique, nous non plus. Néanmoins, il faudra rapidement analyser comment sera géré ce surcroît colossal de dette. Le contexte inédit et l'adoption par le Sénat de budgets essentiels comme ceux de la justice ou de l'intérieur n'auront pas suffi pour parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Je regrette moi aussi ce nouvel échec, qui entraîne une plus faible survie de nos amendements au cours de la navette parlementaire. Il est vrai que, comme chaque année, il y avait Les députés ont finalement supprimé la contribution exceptionnelle introduite par le Sénat sur les contrats d'assurance. Nous espérons que le Gouvernement a obtenu des garanties suffisantes de la part des assureurs, qui jouent un rôle essentiel dans la crise que nous traversons. À eux aussi de faire preuve de responsabilité La plupart des nouvelles dispositions introduites par le Sénat ont été supprimées. Parmi les dispositions néanmoins retenues, je relève le crédit d'impôt pour les agriculteurs engagés dans la sortie du glyphosate et le maintien du volet national d'Écophyto, défendu par Henri Cabanel. Je salue également le maintien des dispositions relatives au renforcement de l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports, proposées par Nathalie Delattre. Je souhaite néanmoins exprimer une inquiétude de plus en plus forte en ce qui concerne les finances locales. Le rapport publié hier par la Cour des comptes a confirmé ce que l'on pouvait entendre depuis plusieurs mois la crise entraîne une fragilisation financière de certaines collectivités, compensée seulement en partie par le plan de soutien de l'État. Je pense en particulier aux départements et à l'investissement public local, alors que le renouvellement des élus constitue une période charnière. En conclusion, je m'interroge quatre révisions de la loi de finances initiale pour 2020. Rendez-vous dans un an pour analyser l'exécution du budget pour 2021, en espérant que nous parviendrons collectivement à maîtriser la situation sanitaire et ses conséquences sociales et économiques,

L'augmentation de la taxe sur les transactions financières, vous n'en voulez pas. L'encadrement de la rémunération des actionnaires, vous n'en voulez pas davantage. Il en va de même de l'instauration d'une taxe sur le poids des véhicules, et non à partir de 1 800 kilos, qui exclut finalement la grande majorité des véhicules. De nombreuses autres propositions sont malheureusement remises à plus tard, après moult concertations et autres réunions dans les ministères qui retardent la mise en place de mesures décidées par les citoyens, pour les citoyens et pour le climat. C'est le Parlement qui décide ! Alors que nous tentions de vous alerter tout au long du budget, nous vous avons également proposé d'instaurer en échange des aides publiques des contreparties environnementales, des contreparties au maintien de l'emploi ou le non-versement de dividendes. Vous nous rétorquez qu'il ne faut pas contraindre les entreprises, surtout en temps de crise. n'est pas le seul à formuler un tel constat : le Haut Conseil pour le climat critique le plan de relance assez vertement, si je puis dire. D'abord, ce que le Gouvernement nous a vendu comme un effort de sincérisation du budget au regard des objectifs environnementaux est un leurre et le plan de relance n'est pas davantage « vert Vous affirmiez que la majorité des dépenses étaient neutres pour le climat, alors que 70 % d'entre elles s'inscrivent dans la continuité et le déni des exigences climatiques. Sur ce point, le Conseil d'État, qui a récemment mis en demeure le Gouvernement, a été également précurseur. Ensuite, le plan de relance ne soutient que marginalement l'emploi et la formation, notamment celle qui est tournée vers la transition bas-carbone, alors qu'elle est fondamentale pour opérer un réel changement de paradigme. Pour finir sur ce sujet, il y a un risque que certaines mesures du plan de relance accroissent encore les inégalités et, par conséquent, les tensions sociales. À défaut d'avoir pu infléchir vos positions sur ces sujets, nous sommes résolus, comme le préconise le Haut Conseil pour le climat, à évaluer les impacts de la politique climatique du plan de relance au regard de différentes dimensions, économique, sociale et politique. lieu de vous appuyer sur les collectivités locales pour affronter la crise sanitaire et mener la relance, vous refusez de restaurer leurs marges de manoeuvre. Ces carences nuiront à long terme à l'investissement public local, qui représente néanmoins encore 70 % de l'investissement public dans notre pays. pays. La Cour des comptes estime, dans son rapport rendu public hier, que, « dans ces conditions, les possibilités de contribution des départements au plan de relance apparaissent plus qu'incertaines ». un constat encore pire : ils vont être incapables d'assumer la hausse des dépenses sociales causée par la précarisation de bon nombre de nos concitoyens dans cette crise. Nous vous l'avons dit, ils devront assumer les dépenses exceptionnelles, parce que l'État n'a pas voulu mener une action différente à l'endroit des plus démunis, des plus éloignés de l'emploi. Leur épargne globale devrait baisser de 45 % en 2020, selon la Cour des comptes. Le Gouvernement ne propose que des mesurettes permettant un sursis en attendant que la bombe à retardement que constituent les avances remboursables ne finisse par exploser. C'est donc un budget quelque peu traditionnel, avec des mesures insuffisantes pour faire face à une crise que les citoyennes et les citoyens traversent très difficilement. Les jours qui viennent s'annoncent sombres, car vous vous cramponnez à vos certitudes sans prendre en compte la profondeur de la crise économique et sociale qui touche notre pays. La parole est à Mme

lois de finances (LOLF) en 2001, nous avons coutume de dire, sans doute à raison, que l'examen du budget par le Parlement se déroule dans des délais très contraints. Une chose est sûre : même en cette période de très grande incertitude, 2020 n'y a pas fait exception. L'exception, cette année, tient au fait que, malgré ces délais d'examen très contraints, le texte a subi des changements majeurs au cours de la navette parlementaire. Cela a été moins dû à nos initiatives parlementaires qu'aux ajustements rendus nécessaires par les évolutions du contexte sanitaire.

Cette modification de l'article liminaire, si elle n'a pas entravé nos débats, a toutefois placé ceux-ci sous le signe d'une instabilité peu propice à la prise de décisions éclairées. Cet ajustement, comme bien d'autres, reflète les fluctuations importantes du contexte macroéconomique. Il prend aussi acte des adaptations stratégiques opérées par le Gouvernement, qui a dû contraindre de nombreux secteurs à maintenir les restrictions sanitaires en cette fin d'année et pour le début de l'année prochaine. En tout état de cause, ce qui compte, c'est non pas tant d'ajuster fréquemment les textes budgétaires que de rester cohérents dans notre politique de soutien à l'économie. En effet, toutes les décisions que nous prenons doivent s'inscrire dans la continuité des décisions déjà prises et de la promesse de soutien que le Gouvernement, avec l'appui du Parlement, a faite à toutes nos entreprises. Cela vaut tout particulièrement pour nos commerçants, nos restaurateurs, nos hôteliers et les acteurs du monde de la culture. Comme des quatre lois de finances rectificatives l'ont déjà montré, le Sénat a su faire preuve d'esprit de responsabilité pour soutenir les dispositifs d'urgence et de soutien. Aussi, le désaccord en commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances a davantage tenu à des choix de stratégie fiscale et budgétaire qu'à des divergences de vues sur les mécanismes de soutien.

Cela vaut notamment pour le financement des collectivités territoriales, au sujet duquel certaines des propositions du rapporteur général, notamment sur les compensations, ont été fort heureusement retenues. C'est aussi le cas pour certains dispositifs de soutien aux entreprises que nous avons améliorés.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre amendement « Coluche » adopté en première lecture a légitimement fait parler de lui, et je m'en félicite. En 1986, Coluche disait déjà : « Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. » Ce budget pour 2021 ne risque pas d'inverser la tendance ... Alors que notre pays et le reste du monde traversent une crise sanitaire sans précédent, nous devons faire face à l'aggravation de la crise sociale et à l'explosion de la pauvreté. Dans un contexte aussi grave, les socialistes regrettent l'absence de toute écoute de la part d'un gouvernement qui n'entend que lui-même. Ces dernières semaines, alors que, dans cet hémicycle, deux visions de droite s'affrontaient, nous portions une voix de gauche, celle d'une alternance possible et crédible. de finances accentue les souffrances des plus précaires et ne permet pas de soutenir notre économie correctement. Au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, nous avons défini une opposition cohérente et responsable pour les finances publiques et nous avons avant tout proposé un budget créant de nouvelles solidarités, soutenant les plus précaires, et réellement écologique. Nous n'avons pas à rougir de nos amendements. Durant ces 145 heures de débat public, nous avons défendu une alternative sérieuse, à la hauteur des enjeux pour notre pays et ses habitants. La jeunesse, frange de la population la plus touchée par la pauvreté, est la grande oubliée de ce budget. Comment cependant oublier l'avenir de notre société ? Notre jeunesse n'a jamais été aussi fragilisée. Monsieur le ministre, ce n'est pas juste « dur d'avoir 20 ans en 2020 », c'est une lutte quotidienne. Nos jeunes sont privés de moyens pour se nourrir, se soigner, étudier correctement ; leurs perspectives se heurtent à la réalité des fins de mois, voire des fins de semaine. Comment penser à l'avenir quand le présent est incertain ? La politique du Gouvernement laisse nos jeunes sombrer dans la pauvreté. En 2019, déjà un quart des jeunes de 18 à 30 ans vivaient sous le seuil de pauvreté. Après cette crise, combien seront-ils ? Au groupe socialiste, nous avons proposé une dotation d'autonomie pour la jeunesse destinée aux jeunes de 18 à 25 ans, la prise en charge élargie des frais de scolarité et d'alternance, ainsi que le financement des projets associatifs ou professionnels. Ces trois mesures pourraient être financées par le seul rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes Il n'y a pas que les jeunes qui subissent la crise sociale de plein fouet, le nombre des inscriptions au RSA a bondi cette année ! Près de 2 millions de foyers ont dû recourir à cette prestation Pour faire face à cette recrudescence de précarité, notre groupe proposait d'autres mesures fortes : une expérimentation du revenu de base, la hausse du RSA, une augmentation de l'aide alimentaire à hauteur de 1 milliard d'euros et la création d'un fonds d'aide au paiement des quittances de loyer. Ces dépenses sont nécessaires et nous devons rester solidaires vis-à-vis des plus démunis. J'entends déjà la petite musique selon laquelle les socialistes videraient les caisses de l'État ... Or nous proposions de financer ces dépenses, non pas par de la dette supplémentaire, mais par des recettes évaluées et chiffrées, qui n'auraient à aucun moment été confiscatoires, comme j'ai pu l'entendre au fil des débats. La politique, c'est faire des choix. De toute évidence, le Gouvernement et la majorité sénatoriale font bien souvent les mêmes, au détriment des plus précaires. Oh ... À titre d'exemple, si nos amendements sur le report des baisses d'impôts pour les entreprises ou sur la sur la suppression de la taxe d'habitation avaient été votés, nous aurions pu financer toutes ces mesures de solidarité ! Je veux également le dire devant vous avec gravité, mes chers collègues : ces recettes supprimées sont aussi celles de nos communes et de nos départements. En effet, les collectivités territoriales n'ont pas non plus été épargnées par ce projet de loi de finances. Le Sénat a d'ailleurs voté un amendement tendant à instaurer un filet de sécurité pour les collectivités, que le Gouvernement a rejeté, mais réintroduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale ! Était-ce trop difficile d'accepter une mesure sénatoriale ? Par ce budget, le Gouvernement affirme son jacobinisme en niant la pertinence même de l'action publique territoriale. Par ailleurs, il faut bien dire que la réorganisation territoriale des services de l'État n'aide en rien. Je pense en particulier publiques. Comme de nombreux collègues ici, je déplore que, avec les fermetures de trésoreries- par exemple dans mon département de la Haute-Vienne -, le redéploiement des services fiscaux ne permette plus d'assurer les missions de conseil auprès des communes et de la population, alors même que celles-ci devaient être maintenues. Il ne faut pas s'étonner du fossé qui se creuse entre le citoyen et les politiques publiques ! En définitive, si la période n'est certes pas facile, le Gouvernement a fait des choix au profit des plus aisés et au détriment des plus modestes.

Il faut bien dire que les propositions des sénateurs n'intéressent guère l'exécutif, qui préfère supprimer presque tous les ajouts du Sénat, quitte parfois à ajouter en nouvelle lecture des amendements quasi identiques à ceux qui ont pourtant été refusés dans cet hémicycle. Ce qui manquait

En responsabilité, nous sommes pourtant parvenus à trouver un accord sur les quatre projets de loi de finances rectificative de l'année 2020, ce qui prouve l'esprit constructif dans lequel travaille le Sénat. Il paraissait pour le moins compromis d'y parvenir sur le projet de loi de finances, dont 285 articles restaient en discussion. Nous regrettons toutefois que l'Assemblée nationale ait si peu tenu compte des votes du Sénat lors de la nouvelle lecture. Comme disait Charles Trenet, « que reste-t-il de ces beaux jours » que nous avons passés à travailler sur le budget avec vous, monsieur le ministre, ce dont je vous remercie, ce dont nous vous remercions

En dehors d'amendements du groupe sénatorial de La République En Marche, qui sont en vérité d'origine gouvernementale- nous le savons tous, car nous l'avons fait avant vous -, et de l'amendement sur le jour de carence défendu par Jean-François Husson avec le Gouvernement, je note que très peu de mesures significatives votées par le Sénat seront retenues dans le texte définitif., principale mesure retenue est la garantie pour 2021 des recettes fiscales du bloc communal, en y incluant les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et surtout la CVAE. Le Sénat a tenu à instaurer un mécanisme de compensation des pertes de CVAE pour les départements et le bloc communal en 2021, à hauteur de 1 milliard d'euros : nous nous réjouissons de la reprise de l'esprit de cette mesure. En revanche, les recettes domaniales et les régies municipales en seront exclues. Concernant ces dernières, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser le dispositif que vous avez prévu de faire passer par ordonnance lors d'un prochain conseil des ministres ?

Par ailleurs, nous nous réjouissons que la mesure défendue par Gérard Longuet depuis trois ans sur la fiscalité liée au stockage souterrain des déchets radioactifs ait été adoptée par les députés.

Nous nous félicitons également de la prolongation jusqu'en 2024 du crédit d'impôt pour les productions cinématographiques et audiovisuelles internationales proposée par Laure Darcos. Exception qui confirme la règle, les députés l'ont votée contre l'avis de leur commission des finances et contre l'avis du Gouvernement.,

Leur écho s'est perdu dans la vallée de Bercy pour déclencher une avalanche de crédits cette nuit : 600 millions d'euros de nouveaux crédits pour soutenir des secteurs touchés, comme le sport, la culture, mais aussi les stations de montagne.

mais en l'améliorant selon plusieurs axes. Nous avons dit « oui » à une relance verte, mais sans écologie culpabilisante, avec la suppression du malus sur le poids, le lissage sur cinq ans du malus sur le CO2 proposé par le rapporteur général, le renforcement de la prime à la conversion et des suramortissements pour les poids lourds et les avions neufs moins polluants. Nous avons dit « oui » à une baisse des impôts de production, tout en la renforçant la diminution du plafond de la contribution économique territoriale et tout en apportant des garanties aux collectivités locales. Nous avons dit « oui

Non aux commerçants. Non à la taxation des assurances, qui a pourtant permis à Bruno Le Maire d'aboutir au gel des primes. Non encore à une garantie des pertes d'exploitation, aux chèques restauration, à un fonds de soutien pour les indépendants. Non au photovoltaïque,

Vous rompez cette unité. Dès que la bise fut venue, ce gouvernement cigale nous oblige à crier famine pour nos amendements ! Ce n'est pourtant pas la morale de La Fontaine, qui dit aussi, dans : « Il se Il se faut entraider, c'est la loi de nature ». Vous avez, de nouveau, choisi d'aller seul. Vous assumerez seul. Dans cette fable, faute d'avoir voulu partager, l'âne se fait dévorer par le loup, car le chien ne vient plus à son aide.

avoir dans cette forme de défiance qui risque de s'installer entre les décisions de l'État et le goût d'inachevé que ressentent les élus des territoires, notamment des communes.

démocratique au service du pays. Lorsque le Sénat s'exprime sur un certain nombre de sujets, qu'il s'agisse de politiques sectorielles ou d'ambitions,

des bourgs-centres et des petites communes de quelques poignées d'habitants. Le Gouvernement s'honorerait, avec sa majorité à l'Assemblée nationale, à mieux prendre en compte ces propositions,

Le scrutin est ouvert.

la commission des affaires sociales a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 11 voix pour, 1 voix contre -à la nomination de M. Jean Bassères aux fonctions de directeur général de Pôle emploi.